La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à accélérer le redressement des finances publiques.

rien de grand ne s’est jamais fait sans l’intuition du temps long. En France, on le voit dans tout ce qui structure encore nos territoires et notre économie.

Le développement du réseau ferré dans l’Hexagone a permis l’essor de nos territoires, en reliant les petits villages de nos campagnes aux grandes villes et aux grands ports. Tout ce pan de l’histoire n’aurait jamais été possible

artisanaux. Nous sommes nombreux ici à souhaiter un renforcement de la planification. Il s’agit non pas de faire l’éloge des méthodes soviétiques pour organiser l’économie et la société, mais simplement,

C’est pourquoi je tiens à saluer cette proposition de loi constitutionnelle, qui nous invite à renouer avec le temps long. L’inversion du rapport entre annualité et pluriannualité pourrait constituer une révolution budgétaire que je crois indispensable. À cet égard, j’ai l’honneur d’affirmer faire preuve de constance. En effet,

Les rapporteurs ont expliqué pourquoi ce qui nous apparaissait alors comme nécessaire et salutaire leur semble aujourd’hui superfétatoire et contre productif.

Mais qui peut dire que tout cela a permis de résoudre la crise budgétaire ? Qui peut dire que la situation s’est globalement améliorée depuis 2011 ? Nos rapporteurs sont ils bien certains que la situation de nos finances publiques n’aurait pas été meilleure si le projet de loi constitutionnelle avait été finalement promulgué ? où nous en sommes si la programmation des finances publiques avait été ainsi renforcée ? Mes chers collègues de la majorité sénatoriale, nous souhaitons tous le rétablissement de nos comptes publics. Bien sûr, il est sain, et même nécessaire, que nous débattions des moyens d’atteindre cet objectif. Nous le ferons longuement à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2025. Mais il est aussi indispensable de changer la méthode par laquelle nous votons le budget, et donc de réviser

agir aussi pour garantir la soutenabilité de la dette publique pour les prochaines générations. Certes, notre action au service du redressement des finances publiques se traduit déjà,

Les grands principes budgétaires qui font la force du modèle français sont aujourd’hui mis à l’épreuve. Il nous incombe, en conséquence, de proposer un cadre plus performant et plus lisible.

de redonner tout son sens au « chaînage vertueux ». Il faut enfin introduire une véritable logique de pluriannualité transversale, au moment où l’on parle beaucoup de planification et de la nécessité d’assurer un contrôle plus strict de nos trajectoires,

financier. Une loi portant cadre financier pluriannuel remplacerait les actuelles orientations pluriannuelles des finances publiques définies dans la loi de programmation des finances publiques.

La solution défendue dans ce texte vise donc à défendre un objectif à la pertinence renouvelée. Toutefois, elle se heurte ce faisant à des obstacles juridiques et pratiques d’importance. En premier lieu, cette solution présente un risque de rigidification excessive du pilotage budgétaire, en particulier de l’action parlementaire en la matière.

Cela reviendrait à remettre en cause le principe constitutionnel d’annualité budgétaire, pourtant essentiel à l’expression du consentement démocratique à l’impôt et au contrôle de l’utilisation de ce dernier. Les droits du Parlement s’en trouveraient nécessairement endommagés.

modalités. Ce risque de paralysie institutionnalisée me semble aller à l’encontre de l’esprit de nos institutions. Le basculement de la fiscalité dans le domaine réservé des lois de finances contribuerait également à amoindrir amoindrir le pouvoir budgétaire du Parlement et, de manière plus large, la capacité d’initiative des parlementaires dans ce domaine. En deuxième lieu, la solution proposée serait susceptible d’entraver la libre administration et l’autonomie financière de nos collectivités territoriales. Ainsi, la fixation pour cinq ans dans une loi cadre de la trajectoire des prélèvements obligatoires aurait nécessairement un effet par ricochet et de long terme sur les ressources des collectivités. enfin, le renforcement du rôle du Conseil constitutionnel et la constitutionnalisation de celui du Haut Conseil des finances publiques suscitent En chargeant explicitement le Conseil constitutionnel d’une mission d’évaluation de la conformité des lois de finances au cadre financier pluriannuel, de loi constitutionnelle risque de transformer en partie l’office du juge constitutionnel : ce dernier deviendrait en quelque sorte un juge financier, exerçant un quasi contrôle d’opportunité sur les décisions, au regard d’indicateurs chiffrés complexes, essentiellement étrangers au droit constitutionnel et remontant parfois à plusieurs années. Cela pourrait contribuer à dénaturer le rôle de cette institution. La décision en matière budgétaire est en effet avant tout de nature politique ; elle doit donc revenir au Parlement et au Gouvernement. compte tenu de la présence de la Cour des comptes dans la Constitution, l’inscription du Haut Conseil des finances publiques n’apparaît pas indispensable. Pour conclure, je rappellerai que la rigidité des procédures n’est pas synonyme de rigueur dans la gestion des affaires publiques.

institutionnels et juridiques. Je partage donc l’analyse prudente du rapporteur pour avis. Néanmoins, nous devons poursuivre notre réflexion sur ce sujet. Les propositions formulées par la commission sur l’avenir des finances publiques qu’a présidée Jean Arthuis apparaissent à cet égard très opportunes, tout en permettant d’agir à cadre constitutionnel constant.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle que nous examinons aujourd’hui soulève des questions fondamentales sur la gestion de nos finances publiques, à un moment où notre déficit atteint des niveaux alarmants. Plus précisément, ce texte a pour but d’inscrire dans la Constitution la primauté d’un cadre budgétaire pluriannuel sur le principe d’annualité. Depuis 1974, aucun budget n’a en effet été voté à l’équilibre et la dette publique s’élève désormais à plus de 113 % du PIB. Ce texte vise donc à instaurer des lois cadres financières pluriannuelles, qui fixeraient pour chaque législature des plafonds de charges et des objectifs budgétaires contraignants dans les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Ses auteurs proposent aussi d’attribuer le monopole des dispositions fiscales aux lois de finances et de constitutionnaliser le Haut Conseil des finances publiques en élargissant ses missions.

sur l’autonomie des collectivités territoriales. La remise en cause du principe d’annualité budgétaire paraît particulièrement problématique. Ce principe, garant du consentement à l’impôt et du contrôle régulier des dépenses, permet au Parlement d’adapter chaque année les budgets aux réalités économiques. L’imposer sur toute une législature risquerait de rigidifier notre cadre budgétaire, compromettant ainsi notre réactivité en cas de crise. De plus, la rigidité de la loi cadre que ce texte propose en Congrès, soulève des questions démocratiques. Cette majorité qualifiée, habituellement réservée aux réformes d’ampleur dépassant les enjeux partisans,

imposer des plafonds de prélèvements obligatoires et des orientations d’investissement centralisées pourrait compromettre leur libre administration financière. Enfin, la constitutionnalisation de critères budgétaires évolutifs imposés par des règles européennes régulièrement révisées pourrait contraindre notre cadre budgétaire de façon disproportionnée. Le Conseil constitutionnel serait chargé de juger la conformité de ces critères en fonction de prévisions, un rôle délicat qui pourrait mettre en péril la cohérence de notre politique budgétaire. Si le groupe RDPI partage l’objectif d’un redressement des finances publiques, nous restons convaincus que c’est avant tout par une volonté politique que nous pourrons instaurer et tenir la discipline financière nécessaire à la résorption du déficit des comptes publics. Nous voterons donc contre ce texte, dont nous tenons toutefois à saluer l’ambition louable de maîtrise des déficits.

loi constitutionnelle que nous examinons vise à inscrire dans notre norme fondamentale le principe de pluriannualité budgétaire, qui prévaudrait sur l’actuel principe d’annualité. Les motivations avancées par l’auteure du texte sont tout à fait louables et ne devraient pas faire l’objet d’une contestation large dans notre assemblée, particulièrement dans le contexte que nous connaissons. S’il n’y a pas lieu d’entrer dans les détails de cette situation, je tiens à souligner que l’instabilité politique participe de ce phénomène qui plonge le monde économique dans l’incertitude.

là avant tout d’un problème politique auquel le droit constitutionnel ne saurait apporter une réponse satisfaisante. Le principe d’annualité budgétaire peut paraître désuet, mais il garantit le contrôle parlementaire du budget, impératif démocratique issu de la Révolution française. La délibération parlementaire annuelle permet à la fois aux citoyens de constater le projet défendu par leurs représentants et au Gouvernement de soumettre sa vision à l’épreuve de la représentation nationale.

le principe d’annualité n’est pas incompatible avec les exigences de programmation imposées par le droit européen et le rythme économique. Il doit au contraire être associé à une surveillance accrue de ladite programmation, comme le préconise le rapport de la Cour des comptes

Le texte prévoit de plus une procédure de révision des lois cadres bien trop stricte, dont la mise en œuvre semble quasi impossible. Si la programmation doit être un guide sérieux et réaliste dans la préparation du budget, elle ne peut devenir un carcan qui rendrait nos discussions actuelles accessoires.

En définitive, ce texte apporte une pierre supplémentaire au débat légitime et nécessaire relatif à nos finances publiques et à la meilleure manière d’en assurer la soutenabilité.

intervient au moment même où la droite tend à imposer une nouvelle austérité sans majorité à l’Assemblée nationale. Enfin, cette proposition de loi constitutionnelle laisse à penser que le Parlement serait responsable de la dette publique. Nous savons tous ici que ce n’est pas vrai.

nous espérons une opposition la plus large possible à cette tentative de rationaliser le Parlement, et partant, de nous contraindre à une démission démocratique. Ce texte portera un coup fatal au débat démocratique, pourtant déjà bien limité. Constitution, qui rend irrecevable toute proposition de financement d’un service public ; l’article 47 1, instauré en 1996 pour cadenasser la démocratie sociale

Ces baisses d’impôt se retrouvent d’ailleurs à l’euro près dans les déficits publics. Pour sa part, le groupe CRCE K prône la planification comme mode de gouvernance budgétaire, non pas pour introduire des rigidités et annihiler le débat parlementaire, mais pour proposer une orientation politique claire, conforme aux besoins de la Nation et non centrée sur les besoins des marchés financiers.

Le Gouvernement décide de ce qu’il faut dépenser, et le Parlement se borne à en prendre acte. Nous gardons notre cohérence, mes chers collègues. Le peuple français n’est pas irresponsable

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’une proposition de loi présentée par notre collègue Vanina Paoli Gagin visant à inscrire dans la Constitution un cadre plus strict pour nos débats budgétaires au travers de lois cadres financières pluriannuelles. Cette initiative, inspirée par la tentative de réforme constitutionnelle de 2011, cherche à ancrer dans notre Constitution des plafonds de dépenses pour contraindre notre approche des finances publiques, dans l’espoir

de choix politiques assumés et, ces dernières années, souvent imposés au Parlement l’activation de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. La méthode proposée aujourd’hui n’est pas la garantie d’un redressement vertueux. pourrait en revanche entraîner des effets de bord délétères, sur les plans tant budgétaire que démocratique. Ce texte porte en lui la réduction de la capacité de l’État et du Parlement à répondre aux défis socio économiques et environnementaux. Cette nouvelle rigidité introduite dans l’élaboration du budget pour notre démocratie et pour notre politique économique. Si la pluriannualité budgétaire est un cadre sécurisant qui peut être promu, notamment dans le respect des lois de programmation, elle doit aussi permettre une certaine flexibilité, notamment en cas de crise. En 2020, face à la pandémie de covid 19, la France a déployé des moyens financiers massifs pour protéger l’économie et les citoyens, montrant ainsi la nécessité de pouvoir intervenir rapidement sans entraves excessives. La règle pluriannuelle stricte prévue par ce texte, en dépit de ce qu’affirme à tort l’exposé des motifs, aveugle aux circonstances, interdit des écarts budgétaires trop importants, puisque ceux ci devront être obligatoirement rattrapés à un rythme peu soutenable.

ancrerait dans la Constitution une règle d’or qui s’imposerait à toutes nos politiques. Une telle révolution copernicienne n’arrive pas en tête des préoccupations de nos concitoyens, contrairement à l’affaissement généralisé des services publics ou aux besoins de base que sont se loger, se nourrir dignement ou vivre en sécurité dans un environnement sain. Bien que cette proposition parte du constat, partagé dans cet hémicycle, de la dégradation continue de nos comptes publics, je rappelle que des baisses d’impôt et des exonérations de cotisations ont largement été votées sur les travées de la majorité sénatoriale. La dégradation des finances publiques est le fruit de choix politiques dont certains ont été soutenus

invoquant la nécessité de « changer la méthode par laquelle on élabore le budget » pour « reprendre la maîtrise de nos comptes », cette proposition de loi constitutionnelle, déposée par notre collègue Vanina Paoli Gagin, vise à modifier ou à compléter les dispositions budgétaires et financières

le monopole des dispositions relatives aux prélèvements obligatoires. Enfin, elle constitutionnalise l’existence du Haut Conseil des finances publiques aux côtés de la Cour des comptes, institution auprès de laquelle le Haut Ce texte s’inspire d’un projet de loi constitutionnelle, déposé en 2011 dans un contexte de crise de la dette souveraine dans la zone euro, qui n’a finalement jamais été soumis au référendum ni au Congrès. Une décision du Conseil constitutionnel disposant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la Constitution pour transposer les exigences européennes a temporairement clos ce débat. Face à la situation dégradée que nous connaissons, il est légitime de nous interroger de nouveau sur la pertinence d’une modification de notre loi fondamentale pour atteindre nos objectifs.

Aujourd’hui, comme en 2008 ou en 2020, la dégradation massive et soudaine des finances publiques résulte d’une crise – celle des en 2008, celle de la covid 19 en 2020 –, mais pas uniquement : les choix budgétaires et fiscaux des gouvernements d’hier et d’aujourd’hui, privant l’État de dizaines de milliards d’euros de recettes, ont largement contribué à alourdir la charge de la dette. Pour le dire clairement, je ne suis pas convaincu que ce texte aurait empêché la dégradation récente de nos finances publiques. La responsabilité première dans cette dégradation est à chercher, me semble t il, du côté de ceux qui écrivent le budget, à savoir le Gouvernement. On pourrait évidemment incriminer ceux qui le votent et l’amendent,

Avec l’instauration de lois cadres pluriannuelles, ce sont bien les marges de manœuvre financières du législateur, déjà faibles, qui seraient encore amoindries. Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale devraient en effet nécessairement s’inscrire dans le cadre pluriannuel qui aura été déterminé en début de législature.

La loi cadre pluriannuelle, dans son principe même, paraît particulièrement inadaptée aux temps de crise, qui exigent réactivité et adaptabilité. Quand un gouvernement peut aujourd’hui faire adopter dans les meilleurs délais une loi de finances rectificative, il serait désormais contraint de réviser le cadre financier pluriannuel, selon des modalités particulièrement lourdes exigeant la convocation du Congrès,

Le présent amendement vise à constitutionnaliser un bouclier fiscal plafonnant à 50 % le taux individuel global d’imposition directe. Le bouclier fiscal créé en 2006 fut l’occasion pour le Conseil constitutionnel de se référer expressément à la notion, jusqu’alors inédite, de confiscation, et partant, d’amorcer explicitement l’exigence du caractère non confiscatoire de l’impôt.

devrait assumer ses propres dépenses ; je ne vois pas pourquoi les dépenses de sécurité sociale d’aujourd’hui reposeraient en partie sur les générations futures : ce n’est ni sain ni moral. le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle d’or interdisant, à compter de 2030, tout déséquilibre global entre recettes et dépenses dans les lois de financement de la sécurité sociale.

à cet amendement : je pense qu’une règle d’or pourrait être instaurée pour les comptes de la sécurité sociale, puisque ce sont effectivement des dépenses courantes, de fonctionnement, et qu’il est anormal

Pour répondre à mon collègue Savoldelli, que j’apprécie particulièrement même s’il nous arrive d’avoir des divergences, il ne s’agit pas de manager de la même façon dans le privé et dans le public.

Mes chers collègues, je vous rappelle que, si l’article 12 n’était pas adopté, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle, dans la mesure où les douze articles qui la composent auraient été rejetés. Aucune explication de vote sur l’ensemble

Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Pour rappel, les Houthis sont un mouvement politique et militaire fondé dans les années 1990. À l’origine, suivant la mouvance chiite, ils avaient principalement des revendications religieuses. Ils s’opposaient également à l’influence étrangère au Yémen, visant en particulier l’Arabie saoudite et les États Unis. C’est en 2014 qu’ils sont devenus un acteur majeur au Yémen et dans la région, après avoir pris le contrôle de la capitale, Sanaa, et contraint le gouvernement yéménite à fuir au sud du pays. Les Houthis, soutenus par l’Iran, contrôlent aujourd’hui une grande partie du Yémen, notamment le littoral donnant sur la mer Rouge. La situation qui s’y présente actuellement dépasse le simple cadre régional ; elle a des implications multiples et profondes, à la fois économiques, écologiques et sécuritaires. La mer Rouge est une voie de passage essentielle par laquelle transite plus de 10 % du transport maritime international. Chaque année, elle voit circuler 25 % du trafic mondial de porte conteneurs. C’est une voie particulièrement stratégique, sachant que plus de 90 % du commerce international en volume passe par la mer. Elle est traversée par des navires qui transportent des marchandises diverses et du pétrole, acheminés vers plusieurs continents, comme l’Europe et l’Asie, dont environ 40 % des échanges transitent par cette voie. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, en octobre 2023, les Houthis ont mené plusieurs attaques contre Israël et contre des navires qui lui seraient liés au large du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Mais pas uniquement ; il s’avère que le terrorisme maritime des Houthis a également un objectif économique. Selon une enquête menée au nom du comité des sanctions du Conseil de l’ONU sur le Yémen, les Houthis perçoivent des « taxes » d’environ 180 millions de dollars par mois auprès de certaines agences maritimes, en échange du renoncement à attaquer leurs navires commerciaux lors du passage de ceux ci en mer Rouge et dans le golfe d’Aden. Les Houthis utilisent des drones et des missiles pour cibler indistinctement des navires civils et militaires, y compris des navires français. Ces exactions ont souvent causé de lourds dégâts matériels et mettent perpétuellement en danger les femmes et les hommes qui sont présents sur les navires pris pour cible.

Un navire coulé ou capturé par les Houthis entraîne une perte économique liée à la marchandise volée, en moyenne 1 milliard d’euros par bateau, pour les entreprises concernées.

Un cadre de la CMA CGM, que j’ai entendu en audition dans le cadre de mes travaux préparatoires, m’a fait l’état des lieux des répercussions de la situation en mer Rouge sur l’armateur français.

sans oublier le coût de la main d’œuvre et du carburant nécessaires pour faire fonctionner ces bateaux. Au delà de leurs impacts économiques dévastateurs sur le commerce maritime, les agressions des Houthis représentent une menace écologique L’exemple le plus flagrant est celui du naufrage du navire en mars 2024, qui transportait 22 000 tonnes d’engrais chimiques et des centaines de tonnes de carburant. Ces substances se sont déversées dans la mer Rouge, créant une nappe toxique de plusieurs kilomètres de long, avant que le navire ne soit définitivement coulé. Je souhaite rappeler, pour mémoire, la catastrophe provoquée par l’ en 1989, lorsque ce pétrolier déversa plus de 40 000 tonnes de pétrole brut dans les eaux de l’Alaska. Cet événement entraîna l’une des pires marées noires de l’Histoire, ravageant plus de 2 000 kilomètres de côtes, tuant des centaines de milliers d’oiseaux marins, de poissons et d’autres types d’animaux et occasionnant des impacts écologiques durables sur l’environnement. Si les attaques des Houthis continuent, nous risquons de voir se répéter de telles catastrophes à une échelle similaire, mettant en péril les écosystèmes marins sensibles de la mer Rouge. En outre, le détournement du trafic maritime de la mer Rouge jusqu’au cap de Bonne Espérance contribue à polluer davantage cette zone. Plus de navires signifie plus de gaz à effet de serre déversés dans l’atmosphère et plus de pollution marine. Je tiens à rappeler que la France est la première concernée par cette situation. En effet, les côtes de l’île de La Réunion sont longées par les navires. Son port et celui de Mayotte sont pleinement mobilisés pour les accueillir, dans des conditions parfois difficiles. Par ailleurs, l’augmentation du volume du trafic maritime accroît les risques de collisions et, par conséquent, le risque connexe de déversements de pétrole dans des zones marines sensibles, y compris sur le littoral français. Des efforts importants pour assurer la sécurisation du détroit de Bab el Mandeb impliquent de grandes puissances mondiales, dont la France. Dès le mois de décembre 2023, les États Unis ont lancé l’opération Gardien de la prospérité, fondée sur une grande coalition de sécurisation maritime, dont la France est partie prenante. Après avoir envoyé la frégate, la France a également rejoint l’opération Aspides. créée en février 2024 par l’Union européenne, vise aussi à répondre aux agressions houthies à l’encontre des navires commerciaux qui transitent par la mer Rouge. Les frégates européennes sont mobilisées quotidiennement pour protéger les rares navires transitant encore par cette zone, qui n’est toujours pas assez sécurisée pour permettre une reprise du trafic maritime mondial. Au delà de ce trafic, c’est notre sécurité à tous qui est en jeu, car la situation actuelle en mer Rouge a des implications et des conséquences qui la dépassent. Depuis 2015, les Houthis dirigent le nord du Yémen, alors que le gouvernement yéménite, internationalement reconnu, s’est réfugié au sud du pays. Comme je l’ai mentionné précédemment, les rebelles ont commencé à attaquer des navires commerciaux après les événements du 7 octobre 2023, prétendant agir par solidarité avec le peuple palestinien. Soutenus par l’Iran, ils affirment être les seuls acteurs au Yémen à opérer au profit de la cause palestinienne. Cherchant à discréditer le gouvernement yéménite et à s’en prendre aux soutiens réels ou supposés d’Israël, les Houthis sont en réalité un atout pour « l’axe de la résistance ». Ils font le jeu de la stratégie régionale iranienne contre l’État Téhéran joue un rôle déterminant dans le renforcement des capacités militaires des Houthis. Ces derniers ont acquis un arsenal sophistiqué, comprenant des missiles balistiques et des drones capables de cibler des infrastructures stratégiques. Il est évident que la situation en mer Rouge est intrinsèquement liée au conflit israélo palestinien. L’implication de l’Iran dans ce conflit fait de cette zone un terrain d’affrontement indirect entre la République islamique et Israël. début d’octobre, nous avons appris que l’Iran servait d’intermédiaire dans des négociations ouvertes en vue de livrer des missiles antinavires supersoniques russes aux rebelles houthis. Le conflit en mer Rouge va donc bien au delà de son ancrage territorial immédiat, au vu notamment de cette implication de la Russie, qui essaie de renforcer ses alliés face aux Occidentaux soutenant l’Ukraine. Chaque attaque houthie est ainsi à réinscrire dans un contexte plus large, dont les répercussions affectent des millions de personnes dans toute la région et au delà. Je fais écho aux propos qu’a tenus le Président de la République lors de sa dernière intervention à l’Assemblée générale des Nations unies. Bien qu’il n’ait pas directement évoqué la situation en mer Rouge, sa volonté de trouver une solution diplomatique au conflit israélo palestinien résonne profondément avec ce que nous y observons. Emmanuel Macron a rappelé que la recherche de la paix et d’une solution diplomatique est le seul chemin viable pour mettre fin au conflit. Il est de notre responsabilité de suivre cette boussole pour désamorcer la crise en mer Rouge et éviter l’escalade. Mes chers collègues, les actions des Houthis sont intolérables : elles mettent en péril des vies humaines ; elles déstabilisent notre industrie maritime ; elles menacent des écosystèmes vitaux ; elles mettent en danger la stabilité internationale.

C’est pour réaffirmer la position de notre pays et sa détermination à poursuivre ses efforts diplomatiques que j’espère, mes chers collègues, que le Sénat adoptera à l’unanimité cette proposition de résolution. La parole

Grand. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, par son soutien, Téhéran a vassalisé le mouvement insurrectionnel des Houthis. Engagés dans une guerre civile au Yémen, ces rebelles servent également les intérêts de l’Iran et de ses alliés. C’est ainsi qu’ils ont participé à des attaques visant Israël. Les Houthis entreprennent également de porter atteinte à la liberté de navigation en mer Rouge, afin notamment de perturber le commerce international. Comme les gardiens de la révolution avant eux, ils se livrent à des actes de piraterie à des fins de rançon, quand ils ne détruisent pas tout simplement leur cible. Ni la France ni la communauté internationale ne peuvent les laisser faire ! Hélas ! ces attaques entraînent parfois la mort de membres d’équipage des navires marchands. Nous pensons à ceux qui sont tombés, ainsi qu’à leur famille.

12 % du commerce international passait en effet par la mer Rouge, entre le canal de Suez et le détroit de Bab el Mandeb. Or, depuis le début des attaques, le trafic y a chuté de 20 %.

Depuis plusieurs mois, les femmes et les hommes de la Marine nationale tentent de préserver la liberté de navigation en mer Rouge. Sous le feu des rebelles houthis, ils protègent les navires contre leurs attaques ; ils détruisent leurs drones et leurs missiles balistiques. situation démontre l’engagement et les capacités de nos armées, qu’il convient de saluer. Elle renforce également notre conviction que leurs moyens doivent encore être augmentés. Les Houthis ont annoncé vouloir étendre leurs opérations à l’océan Indien. Nous devons souhaiter qu’ils n’y parviennent pas, mais nous devons surtout nous donner les moyens de les entraver. Voilà plusieurs années que nos marins nous signalent une montée généralisée

Dans ce contexte tendu, nous devons veiller à doter nos armées des moyens suffisants pour défendre la France et ses intérêts, mais aussi pour lui permettre d’apporter son concours aux opérations internationales de sécurité – cela passera, naturellement, par les débats que nous aurons dans

trinque, puisqu’il se trouve dans une situation humanitaire déplorable. Seule une authentique voie fédérale permettrait au Yémen de se stabiliser, mais cela supposerait aussi que les États voisins de la région renoncent à instrumentaliser tel ou tel acteur de la scène politique yéménite.

Cette attaque et la pollution qu’elle a engendrée ont eu un impact évident, non seulement sur l’écosystème marin du détroit, mais aussi, évidemment, sur les communautés de la côte yéménite, dont beaucoup dépendent de la pêche. D’autres attaques ont également touché deux villes égyptiennes en octobre 2023, faisant six blessés. Enfin, de nombreux missiles ont ciblé Israël, faisant un mort et plusieurs blessés à Tel Aviv, en juillet dernier. Ces attaques ont mis le Yémen, l’un des berceaux de notre civilisation, sur le devant de la scène internationale. Je souhaiterais attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que ce conflit en mer Rouge s’inscrit dans une histoire plus large, celle du Yémen et celle du sud de la péninsule arabique dans son ensemble.

Dix ans plus tard, en septembre 2014, les Houthis, toujours en conflit avec le gouvernement, ont lancé une insurrection qui a scindé le pays en deux, et qui a contraint les autorités officielles à se retrancher dans le nord est du pays, abandonnant d’ailleurs la capitale, Sanaa. Ce conflit, marqué par de très nombreuses interventions d’acteurs régionaux, dont l’Arabie saoudite et l’Iran, a provoqué l’une des plus graves famines que le monde ait connues depuis un siècle, selon les Nations unies. En effet, comme souvent, ce sont les civils qui paient le prix fort de ce terrible conflit. Les enfants, tout particulièrement, vivent un cauchemar depuis que la guerre civile a éclaté en 2014 : 5 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition au Yémen, ainsi que 1,3 million de femmes enceintes et allaitantes. 70 % de la population a besoin de l’aide humanitaire. Au total, l’ONU estime que plus de 11 000 enfants ont été tués ou gravement blessés, quand 4 000 d’entre eux ont été enrôlés par les milices houthies. Les attaques récentes contre les civils et les navires marchands passant dans le détroit de Bab el Mandeb s’inscrivent dans ce contexte. Leurs conséquences sont connues : 75 % des exportations européennes transitaient par ce détroit avant novembre sept des dix principales compagnies maritimes internationales ont cessé d’emprunter cette route. Depuis février dernier, l’Union européenne a lancé une mission de protection des routes maritimes dans la péninsule, à laquelle la France participe.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la mer Rouge est une voie de passage stratégique pour le transport des marchandises, notamment les produits énergétiques, entre l’Europe, l’Asie et l’Afrique.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a publié le 1 novembre dernier un rapport nous alertant sur le fait que la milice houthie devenait progressivement « une puissante organisation militaire ». La rébellion disposerait désormais de 350 000 combattants, soit dix fois plus qu’il y a dix ans.

Ces attaques mettent en péril la vie de nombreux civils, notamment sur les navires, et constituent une entrave à la liberté de navigation et au droit international. Le 19 février 2024, l’Union européenne a lancé l’opération

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 8 octobre 2023, au lendemain des attaques terroristes du Hamas contre l’État israélien, que nous condamnons fermement, Washington a déployé en Méditerranée orientale un groupe aéronaval visant à dissuader l’Iran de toute intervention directe. Les actes de piraterie des Houthis pour rançonner les navires commerciaux en mer Rouge ont commencé le même jour. Les États Unis ont alors Les États Unis ont alors pris l’initiative de créer une coalition internationale, afin de bombarder, sans mandat, les positions houthies et de protéger les navires commerciaux passant dans ce secteur. L’Union européenne lancera une opération similaire, sous mandat onusien, à l’exception près que cette intervention n’aura pas vocation à bombarder le Yémen. Avec près de 190 attaques depuis la fin de 2023, les Houthis restent aujourd’hui capables de mener de nouveaux assauts.

Comme les auteurs de cette proposition de résolution, nous pensons que chaque conflit armé est un désastre, d’abord humain, mais aussi écologique. Les armes tuent directement, mais aussi indirectement en empoisonnant pour des dizaines, voire des centaines d’années, l’environnement. Par exemple, la sale guerre que mène Poutine en Ukraine a déjà fait plus de 300 000 morts des deux côtés, mais elle a aussi rayé de la carte plus de 100 000 mètres carrés de forêts, qui ont été ravagées par des incendies, et provoqué l’enfouissement dans les sols de milliers de mines remplies de métaux lourds, qui contamineront les nappes phréatiques

je parle des crimes de guerre et du risque plausible de génocide commis en ce moment même, à Gaza, par Netanyahou et son gouvernement d’extrême droite. Il s’agit d’un véritable massacre : des dizaines de milliers de morts et de blessés, des destructions entières de bâtiments,… C’est vrai ! … sur un territoire qui subit déjà,

et soutient des groupes terroristes partout dans la région. Seule une solution politique permettra de faire reculer l’usage de la force, de rétablir la confiance entre les États et de marginaliser les groupes paramilitaires qui gangrènent cette zone. Là encore, la France doit œuvrer à faire entendre sa voix pour imposer un cessez le feu immédiat, contribuer à l’ouverture d’un couloir humanitaire, à la libération des otages détenus par le Hamas et des prisonniers politiques palestiniens, et au respect du droit international en reconnaissant, enfin, l’État de Palestine.

plus de 400 000 morts et près de 200 000 réfugiés. Cette guerre oppose les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, au pouvoir central, appuyé par l’Arabie saoudite et sa coalition. On retrouve, en toile de fond, la rivalité historique entre ces deux puissances régionales. Les superlatifs sont, hélas ! insuffisants pour décrire la catastrophe humanitaire qui accable le Yémen aujourd’hui. Selon l’Unicef, 70 % de la population a besoin d’une aide humanitaire

La jeunesse yéménite n’est pas épargnée : plus de 4,5 millions d’enfants, soit 40 % des enfants du pays, ne vont plus à l’école. Quel avenir envisager pour cette génération ? Comment éviter que le désespoir ne forme le terreau de conflits futurs ? Aujourd’hui, alors que nos intérêts économiques sont touchés, l’attention internationale s’est réveillée. Mais n’oublions pas que, pendant près de dix ans, l’Occident a répondu par un silence assourdissant aux appels de détresse du peuple yéménite. La communauté internationale a une responsabilité

la paix dans la région passera nécessairement par une résolution du conflit israélo palestinien fondée sur le respect mutuel et le droit international. C’est à cette condition que nous pourrons espérer un avenir pacifié pour les peuples du Moyen Orient.

Nous aspirons à une paix véritable, fondée sur le respect et la coopération entre tous les acteurs. Forts de cette conviction, nous apportons notre soutien à cette proposition de résolution, en espérant qu’elle contribue à tracer la voie d’une paix durable. La parole durable. La parole est à Mme Hélène Conway Mouret.

Ce n’est pas la première fois que cette région du monde attire notre attention. La dernière crise de piraterie dans la Corne de l’Afrique, et plus particulièrement dans le golfe d’Aden, remonte aux années 2008 à 2012. Elle découlait principalement de la déstabilisation de la Somalie, État failli s’il en est. À l’époque déjà, une réponse internationale avait été apportée à cette menace contre la libre circulation. En 2008, l’Union européenne a lancé l’opération Atalante, à

c’est l’opération Aspides, engagée en février 2024, dont le mandat est d’intercepter les assauts et d’escorter les navires commerciaux entre le golfe d’Aden et la mer Rouge. Formée sur l’initiative de l’Italie, elle réunit les marines de sept États européens, dont trois ont un bateau présent sur place : la Grèce, l’Italie et la France. Notre pays a fait le choix politique de s’impliquer activement dans cette coalition,

Le détournement du trafic par l’Afrique affecte particulièrement les ports européens de la Méditerranée. L’Italie, dont le commerce dépend à 54 % des voies commerciales maritimes, a perdu 9 milliards d’euros en 2024.

Elle nous permet également de réaffirmer notre position avec force : la France, résolument solidaire de ses partenaires européens et internationaux, continuera de répondre présent pour restaurer la stabilité dans cette région essentielle à l’équilibre mondial.

Elles empêchent les liaisons maritimes avec nos territoires de l’océan Indien, Mayotte et La Réunion, déjà fortement perturbées. Dans ce contexte, le Sénat doit se prononcer sur une proposition de résolution du groupe RDPI condamnant les méfaits des Houthis en mer Rouge et appelant à une action internationale pour protéger le commerce maritime.

Lorsque la coalition menée par l’Arabie saoudite a commencé à lutter contre ces milices, elle a suscité énormément de réactions. Mais vous comprenez bien que l’Arabie saoudite,

Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs,

Cette proposition de résolution s’inscrit dans la pleine continuité de l’action déterminée menée par le Gouvernement pour répondre aux attaques inacceptables perpétrées par les rebelles houthis en mer Rouge. Depuis le début de la guerre à Gaza, ces combattants yéménites insurgés se réclamant de la cause palestinienne multiplient les assauts indiscriminés contre les navires de commerce internationaux battant pavillon au large du Yémen. Soutenus et armés par la République islamique d’Iran, ils portent la responsabilité de plus de 150 actes d’agression depuis le mois de novembre 2023. Ils ont, en outre, visé à de nombreuses reprises le territoire israélien. Cette escalade belliqueuse fait planer une menace croissante sur la sécurité de la région. Dotés de moyens de plus en plus sophistiqués, grâce aux armes venues d’Iran, les Houthis ont franchi un cap supplémentaire dans la violence : le recours aux drones et aux missiles balistiques est devenu une réalité tristement ordinaire. Le sort du cargo britannique , en février dernier, illustre cette montée de la brutalité. Frappé par deux missiles, ce vraquier chargé de 22 000 tonnes d’engrais chimiques a fait naufrage, suscitant de vives inquiétudes environnementales.

Plusieurs marins y ont en effet trouvé la mort. Ces victimes innocentes témoignent de l’horreur et de la gravité de ces assauts, qui font régner la terreur sur les mers. Parce qu’il entrave le commerce international, ce climat de peur porte directement atteinte aux intérêts de la France, ainsi qu’à ceux de l’Europe et de nos partenaires international (FMI) enregistrait une baisse de 30 % du trafic de conteneurs la mer Rouge, tandis que la Commission européenne évoquait une diminution des flux de 22 % dans cette région stratégique. La perturbation des chaînes d’approvisionnement fait pression sur les prix de consommation et risque d’aggraver l’inflation qui pèse sur nos concitoyens. Face à cet engrenage dangereux, la France appelle à l’arrêt immédiat des exactions commises par les Houthis.

équipage. Face à l’ampleur de cette menace, nous ne nous contentons pas d’élever la voix : avec l’appui de nos partenaires européens, nous avons adopté une posture défensive en mer Rouge. Le 19 février dernier, sous l’impulsion de la France, l’Union européenne a donné le coup d’envoi de l’opération maritime Aspides, dont l’objectif est de rétablir la sécurité maritime et de garantir la liberté de navigation au large du Yémen. ce titre sont significatifs : plus de 270 navires ont été escortés. De surcroît, de nombreux drones et missiles lancés par les Houthis ont été interceptés. Cette opération est un témoignage fort de la volonté sans faille de la France et de l’Union européenne de restaurer la sécurité dans cette zone de passage cruciale. Le succès du remorquage du pétrolier, pris pour cible par les Houthis, a notamment permis d’éviter une catastrophe environnementale d’envergure. Cette action coordonnée le confirme : l’Union européenne est déterminée à stabiliser cette région stratégique et à prévenir toute escalade. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, là où le droit international est menacé, la France, fidèle à son héritage et guidée par les idéaux qui la façonnent, s’érigera toujours pour le protéger. La sûreté maritime et la liberté de navigation en mer Rouge, garanties fondamentales des échanges mondiaux et de la sécurité de nos partenaires, traduisent des principes intangibles qui mobilisent toute notre vigilance. À l’unisson des autres nations européennes, la France continuera de veiller sur ces eaux, afin qu’elles deviennent libres et sûres.

sur l’appui indéfectible de ses partenaires et œuvre sous l’égide de l’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, Hans Grundberg, ne reculera devant aucun effort pour ranimer la flamme de la paix au Yémen.

la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Je mets aux voix la proposition de résolution. J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Rassemblement des

des démocrates, progressistes et indépendants, la discussion de la proposition de loi visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans, présentée par Mme Samantha Cazebonne et plusieurs de ses collègues Dans la discussion générale, la parole est à Mme Samantha Cazebonne, auteure de la proposition de loi.

nous nous réunissons aujourd’hui pour aborder une question qui transcende les clivages politiques et les traditions, celle de la protection de nos enfants contre l’exposition à la violence, en particulier à l’occasion de spectacles tels que les corridas et les combats de coqs. Ces pratiques sont reconnues comme des actes de cruauté aux termes de l’article 521 1 du code pénal, mais bénéficient d’une exception pénale lorsqu’une tradition locale est invoquée. Ce motif dérogatoire, d’ordre culturel, ne saurait pour autant atténuer leur caractère cruel et violent. Il est indéniable que, ces dernières années encore, l’État et le législateur ont exprimé la volonté de protéger les mineurs de l’exposition à la violence, en raison de leur vulnérabilité, laquelle a été reconnue par des dispositions légales. aux articles 226 14 et 434 3 du code pénal. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et encadre, quant à elle, la diffusion de la tauromachie à la télévision afin d’éviter de heurter la sensibilité des téléspectateurs, en imposant une signalétique jeunesse et en interdisant la diffusion de la mise à mort.

la mise à mort d’un animal, dont l’incapacité de s’enfuir, cloîtré dans cette arène close, et la compréhension d’une fin proche le rendent agressif envers les hommes à cheval et ceux qui se trouvent dans l’arène. On le fait donc courir dans tous les sens, on le pousse, on le pique, on le harcèle jusqu’à son épuisement. Et la foule qui hurle, massée autour de moi, des “olé” à qui mieux mieux… donc ça, une corrida ? Hurler de manière insensée, fatiguer un animal, jusqu’à lui enfoncer des piques dans son corps meurtri ? C’est donc ça, une fête, pour certaines personnes ? Regarder, jusqu’à être obnubilé, la mort d’un taureau Le taureau s’est effondré sur ses pattes avant, et le coup de grâce est venu, mettant fin à ce carnage. Je n’arrive même pas à trouver un mot plus fort exprimant ma colère, mon impuissance et mon étonnement face à ce spectacle. Tout se mélange, tout le monde hurle de joie, l’animal meurt, et je suis dégoûtée. C’est parce qu’elle était forcée d’assister à cette cruauté que, dans son livre intitulé, Marina Ruiz Picasso évoquait avec franchise les traumatismes

alors que leur compréhension des valeurs de compassion et de bienveillance est encore en pleine formation ? Nous avons le devoir de protéger leur innocence. Par ailleurs, il faut prendre en compte le conflit de loyauté auquel nos enfants peuvent être confrontés. En effet, combien d’entre eux osent dire non lorsqu’ils se trouvent sous l’influence d’un parent enthousiaste et déterminé à l’idée d’assister à une telle atrocité ? Cette pression émotionnelle peut les pousser à participer à des spectacles qui violent les normes fondamentales fondant le respect pour la vie. Les traumatismes résultant de l’exposition à des images de violence ne doivent pas être sous estimés. De nombreuses études documentent leur impact négatif sur le développement moral et comportemental de nos jeunes.

convention doivent rendre des comptes et veiller à ce que toute recommandation soit suivie. L’absence de mention de ces pratiques dans les rapports fournis au Comité témoigne d’une complaisance que nous ne pouvons plus accepter. Mes chers collègues, nous qui ratifions régulièrement des conventions internationales, comment pouvons nous, en toute conscience, ignorer les recommandations de ce comité ? Nous le savons, Nous le savons, en ratifiant une convention, nous nous engageons. Nous ressentons une fierté collective et individuelle chaque fois que les droits des enfants progressent et que nous votons en leur faveur. Alors, pourquoi ne serions nous pas tout aussi fiers de voir d’exposer les enfants à la violence et à la cruauté appliquée sans exception ? Pourquoi une exception existerait elle ici, en France, pays de l’égalité ?

Leur mobilisation est un exemple de courage et de détermination. Mes chers collègues, j’ai suivi avec attention le travail que vous avez effectué au sein de la commission des lois. Celle ci a estimé que « le dispositif proposé était inapplicable en l’état », que le texte « n’apportait pas de solution adaptée au renforcement de la protection des mineurs et était susceptible de poser d’importantes difficultés

La forme devient soudainement primordiale dans l’argumentation de la commission. Pourtant, le recours à des contorsions juridiques pour maintenir un état d’exception permettant d’exposer des enfants à une pratique que nous interdisons partout ailleurs semble paradoxal.

En outre, pourquoi ne pas avoir réfléchi à la question des peines, jugées surdimensionnées ? Pourquoi, si la forme est le problème, monsieur le rapporteur, n’a t il pas été proposé une solution de substitution,

Il n’y est à aucun moment fait mention de la chasse ni d’une quelconque abolition de la corrida. Je fais appel à votre honnêteté intellectuelle, mes chers collègues. Je sais pouvoir compter dessus. En conclusion, il est de notre devoir de refuser toute forme de complaisance face à cette réalité. Nous devons agir avec conviction et voir la réalité en face, sans laisser penser ou dire que cette proposition de loi n’aurait pas lieu d’être, au prétexte que le canal législatif ne serait pas le bon,

Ensemble, faisons en sorte que notre engagement mène à un avenir où les droits des enfants sont respectés sur l’ensemble du territoire national, sans exception. Vous avez excédé votre

la proposition de loi soumise à l’examen du Sénat vise à interdire la présence des mineurs de 16 ans aux courses de taureaux et aux combats de coqs. La commission des lois n’a pas adopté le dispositif proposé, considérant qu’il n’était pas adapté à l’objectif du texte.

il ne semble pas opportun que la loi se substitue aux parents dans le cadre d’un régime juridique reposant sur des traditions locales avérées. La proposition de loi entend couvrir à la fois les combats de coqs et les courses de taureaux.

La pratique traditionnelle des combats de coqs, en particulier dans les outre mer, s’en trouverait fortement affectée, sans qu’il y ait eu de concertation préalable avec les acteurs de terrain. Outre le risque d’un déport vers des pratiques de combats illégaux, il est à craindre que cette mesure soit perçue comme une remise en cause des traditions locales et une source de tensions inutile, surtout dans le contexte actuel. En ce qui concerne les courses de taureaux, je voudrais formuler différentes observations, qui ne relèvent pas de questions de forme. Tout d’abord, la proposition de loi interdirait la présence de mineurs de 16 ans, y compris pour les courses de taureaux sans mise à mort, dès lors qu’il sera considéré que des sévices sont exercés sur des taureaux.

À l’inverse, la proposition de loi ne dit rien des écoles taurines. Si l’effet des mesures proposées est d’interdire aux mineurs de 16 ans de participer aux corridas, la question de l’apprentissage de ces pratiques dans les écoles de tauromachie reste entière.

qui forment à la tauromachie n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte, qui ne vise que les courses de taureaux. Le dispositif proposé interdirait donc aux mineurs de 16 ans d’assister aux corridas, mais permettrait aux parents d’inscrire leurs enfants, dès l’âge de 6 ans ou de 8 ans, dans les quelques écoles de tauromachie que compte notre pays. Plus grave encore du point de vue du droit, la proposition de loi entend traiter la question de la protection des mineurs, en l’insérant dans deux articles du code pénal relatifs au bien être animal. Le texte n’apportant aucune modification au régime pénal, il fait reposer sur l’organisateur la responsabilité liée à la présence d’un mineur de 16 ans.

transformerait, du point de vue pénal, un spectacle légal en sévices graves infligés à un animal, avec plusieurs circonstances aggravantes, dont celle d’avoir commis un acte ayant entraîné la mort de l’animal

J’en viens maintenant à la question de fond : la loi doit elle déterminer, à la place des parents, l’âge auquel il est possible de voir une corrida ?

loi tend à substituer l’appréciation du législateur à celle des collectivités concernées. Or ce choix pose question, étant donné le régime juridique spécifique qui s’applique aux courses de taureaux et aux combats de coqs.

Enfin, la commission des lois a estimé inopportun de substituer l’appréciation du législateur à celle des parents. Eux seuls, dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, elle même encadrée par le code civil et, éventuellement, par le juge aux affaires familiales, déterminent si leurs enfants mineurs peuvent assister ou non à un spectacle fondé sur une tradition reconnue par la loi. Pour toutes ces raisons, sans nier le caractère intrinsèquement violent des spectacles de combats d’animaux, la commission des lois a estimé que

en tant que garde des sceaux, je partage la préoccupation légitime des auteurs de cette proposition de loi relative à la protection des enfants. en particulier du risque de surexposition des mineurs à des images violentes, en direct ou diffusées différents supports de communication. L’intérêt supérieur de l’enfant doit toujours être la boussole qui nous guide. Le ministère de la justice est certes celui qui sanctionne, mais c’est aussi celui qui protège, notamment les plus vulnérables. Toutefois, cet objectif bien légitime de protection des enfants ne doit pas nous faire perdre de vue que les premiers protecteurs de l’intérêt de ceux ci sont ses propres parents. L’autorité parentale est définie par le code civil comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Ses titulaires sont donc, j’y insiste, les premiers gardiens de l’intérêt supérieur de l’enfant : c’est à eux que revient la tâche d’apprécier,

Ainsi, il est de la liberté de chacun de choisir sa culture, ses coutumes, ses pratiques. L’État ne doit pas intervenir, sous peine de se montrer paternaliste, voire invasif, et de déresponsabiliser les parents. À chacun son rôle. Le moyen de la pénalisation, en outre, n’apparaît pas adapté. Va t on pénaliser les parents qui laissent leur enfant regarder des vidéos sur les réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéo violents ? Cela ne viendrait à l’idée de personne, non pas parce que l’intérêt poursuivi n’est pas compréhensible, mais parce que ce n’est pas en sanctionnant pourrons résoudre le problème. Au contraire, on risquerait de braquer, qui plus est lorsque la question est culturelle. Une politique de prévention est bien plus efficace en la matière.

l’abandon, les expériences illicites, les atteintes volontaires et involontaires à la vie de l’animal, ainsi que les mauvais traitements. Nous nous assurons de fixer les orientations et suivons la bonne application de cette politique pénale sur l’ensemble du territoire français.

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

notamment par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 juin 2004, qui a fait date. Ainsi, l’exigence d’une tradition « locale » doit faire l’objet d’une appréciation relativement stricte,

La persistance d’une tradition taurine peut toutefois être déduite de l’intérêt que lui porte un nombre suffisant de personnes, comme l’a décidé la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2006. Une tradition locale ininterrompue permettant la tenue de courses de taureaux a ainsi été reconnue pour certaines communes des régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Sud – Provence Alpes Côte d’Azur. Les territoires concernés par les combats de coqs couvrent une cinquantaine de communes des départements du Nord et du Pas de Calais, mais aussi La La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Polynésie française. C’est bien la preuve du caractère circonscrit du périmètre géographique concerné. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur cette question. Dans une décision du 21 septembre 2012, il a jugé que l’exclusion de responsabilité pénale applicable uniquement dans les parties de territoire national où une tradition ininterrompue est établie ne méconnaissait pas

L’étude attentive de la jurisprudence démontre, de même, que le Conseil constitutionnel a entendu exercer un contrôle sur la nature même de la pratique. À l’occasion de l’examen de l’incrimination de la création de nouveaux gallodromes, prévue au huitième alinéa de l’article 521 1 du code pénal, le juge constitutionnel a déclaré une telle incrimination conforme à la Constitution, considérant que « si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l’exclusion de responsabilité pénale sur l’existence d’une tradition ininterrompue, il s’agit toutefois de pratiques de pratiques distinctes par leur nature ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 susvisée que le législateur a entendu encadrer plus strictement l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces pratiques ; qu’en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ». Là aussi, la jurisprudence est venue encore restreindre le périmètre concerné et trouver un point d’équilibre qu’il serait préjudiciable de venir bousculer. bousculer. La proposition de loi tend à interdire aux mineurs de 16 ans l’accès aux courses de taureaux et aux combats de coqs, alors que le droit en vigueur ne contient aucune restriction d’âge. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit le fait que cette disposition, au delà du bouleversement de l’équilibre jurisprudentiel évoqué, pourrait avoir un effet secondaire important, puisqu’elle sous tendrait un contrôle de l’âge légal des participants, mesure lourde, contraignante, qui n’existe – je le redis – nullement jusqu’à présent et qui n’apparaît pas proportionnée. Cet effet de bord serait d’autant plus marqué que, s’agissant des combats de coqs, l’accès est libre, sans vente de billets. En conclusion, le Gouvernement, s’il partage les préoccupations légitimes liées à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la lutte contre la maltraitance animale, n’estime pas que les dispositions proposées soient à même d’atteindre l’objectif visé. celles ci remettent en question l’équilibre jurisprudentiel et pourraient entraîner des effets de bord non négligeables. C’est pourquoi le Gouvernement est défavorable à l’adoption de cette proposition de loi. La parole

Ce n’est pas anodin, car il s’agit là d’un pan de notre culture que l’on voudrait pouvoir librement transmettre aux jeunes générations. Comme toute culture, elle nécessite que l’on s’y intéresse sans préjugés afin de l’apprécier pleinement

nous ne détournons pas le regard, mais cherchons, autant que possible, à la magnifier. Étrangement, dans une société toujours plus aseptisée et numérisée, où l’on parle de plus en plus de transhumanisme, la corrida et son récit trouvent davantage de sens et nous interrogent sur notre rapport à la mort, et donc à la vie.

que nous examinons aujourd’hui, permet d’aborder des sujets de société qui, malgré les apparences, ne sont pas foncièrement opposés : la protection des mineurs et le respect des traditions culturelles de notre pays. Je sais que beaucoup d’entre vous se positionnent contre l’interdiction de la corrida et des combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans.

Comme l’exposé des motifs de la proposition de loi l’indique, le code pénal comporte de nombreuses dispositions protégeant les mineurs de messages ou d’images, quels qu’ils soient, à caractère violent. les corridas et les combats de coqs peuvent être violents et sanglants, et débouchent généralement sur la mise à mort d’un animal.

Pourquoi ne pas protéger nos enfants de cette violence, alors que le droit français prémunit déjà les mineurs contre une trop grande exposition à la violence virtuelle dans les films ou les jeux vidéo ? Bien que je sois favorable à la mise en cohérence de notre législation, je comprends les réticences de celles et ceux qui craignent que le texte porte atteinte à l’autorité parentale, et surtout à la liberté de chaque parent d’éduquer ses enfants comme il l’entend. La tauromachie et les combats de coqs sont des pratiques profondément ancrées dans le patrimoine culturel français. Il est légitime de vouloir préserver cet héritage ; par conséquent, il est fondé de ne pas chercher à s’ingérer dans le parcours éducatif des familles, et de laisser le choix plein et entier aux parents de transmettre ces traditions à leurs enfants. Je reconnais aussi la complexité soulevée par l’argument de la discrimination. mineurs l’accès aux arènes tout en leur permettant de participer à d’autres activités impliquant la mise à mort d’animaux, comme la chasse, pourrait ainsi être perçu comme une atteinte au principe d’égalité. Cette contradiction mérite notre attention, ne serait ce parce qu’elle pourrait nuire à la crédibilité du texte. D’un point de vue économique, il est indéniable que les écoles de tauromachie et les élevages de taureaux représentent un secteur d’activité qui crée des emplois dans nos territoires. les écoles taurines ne se contentent pas de former de futurs : elles transmettent également des valeurs de discipline, de courage et de respect et participent à l’ancrage culturel de nos territoires. Nous ne pouvons pas ignorer l’impact financier de l’interdiction de la corrida aux mineurs pour ces écoles et pour les passionnés qui, depuis des générations, font vivre cette culture. Cela vaut également pour les combats de coqs,

Cependant, mes chers collègues, il est essentiel de se demander si une tradition peut justifier l’exposition des enfants à des scènes montrant parfois une violence crue. Nos sociétés évoluent, et il est parfois nécessaire de réévaluer certaines pratiques culturelles à l’aune des valeurs que nous défendons aujourd’hui. Encourager l’évolution de nos traditions n’est pas synonyme d’une éradication de notre patrimoine c’est, au contraire, leur offrir une voie de renouvellement et leur permettre de s’inscrire dans la modernité. Cette question délicate nous incite à trouver un équilibre entre la préservation de notre patrimoine culturel et la nécessité de protéger nos mineurs et de favoriser le bien être animal.

Je sais à quel point cette assemblée est attachée à la défense des territoires et de leurs traditions locales, dont la corrida fait incontestablement partie. Ainsi, les fêtes taurines sont devenues des corridas ritualisées à partir du XVI siècle,

Il s’agit non pas d’interdire une tradition, mais de l’encadrer et de la mettre en conformité avec notre sensibilité actuelle, ce qui est singulièrement différent.

Mais, au fond, le sens du dispositif proposé est très simple : modifier le code pénal afin que seules les personnes de plus de 16 ans puissent assister aux spectacles de tauromachie et aux combats de coqs. Pourquoi ? Car assister à ces spectacles, d’une violence certaine et d’une cruauté déjà reconnue par la loi, n’a absolument rien d’anodin.

relève l’absence de logique à vouloir voter un texte sur des pratiques qui concernent uniquement les taureaux et les coqs. Pourquoi ne pas légiférer sur le bien être animal dans son ensemble ? Enfin, l’on cite l’absence de concertation avec les principaux intéressés. Ces arguments ne m’ont pas convaincue. J’y insiste, le seul intérêt de ce texte réside dans une meilleure protection des enfants. Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, les membres du groupe du RDSE voteront, comme à leur habitude, librement sur ce texte, qui aura eu le mérite de nous faire débattre franchement. La parole

3 228 milliards d’euros de dette publique, les ravages du narcotrafic, les enjeux migratoires et écologiques : je pourrais évidemment continuer la liste des défis majeurs qui sont devant nous et qui donnent déjà lieu à des échanges des échanges vifs et animés. Dans une période où le débat public est souvent très tendu, avec une Assemblée nationale morcelée, y avait il urgence à se préoccuper de l’accès des mineurs aux corridas et aux combats de coqs ? Avant d’aborder le fond du débat, je pense qu’il est légitime de se poser cette question. Bravo ! À une très large majorité, notre groupe considère que, non, cela n’est pas le plus urgent et que, oui, cela pourrait raviver des tensions dont nous n’avons pas besoin en ce moment. Ces tensions sont d’autant plus certaines que le débat est en réalité semé de faux semblants. En effet, la cible n’est pas celle qui nous a été présentée par les auteurs de la proposition de loi., le véritable enjeu chacun ici l’a bien compris –, c’est l’interdiction des corridas et des combats de coqs, moins par souci de protection des mineurs que pour défendre une certaine vision de la condition animale. Cette position peut être défendue par certains

nous ne saurions appliquer un dispositif pénal identique aux corridas et aux combats de coqs, dans la mesure où ces activités présentent des différences non seulement pratiques, mais aussi territoriales et culturelles. Par exemple, si l’extinction du combat de coqs représente un objectif pour le législateur, les courses de taureaux font l’objet d’un régime moins restrictif – en témoigne la possibilité de construire de nouvelles infrastructures taurines.

En outre, il s’agit généralement de manifestations en libre accès, souvent associées à des paris. En contrôler l’accès serait coûteux et difficile alors même que nous ne disposons d’aucune certitude quant à l’intérêt d’un tel dispositif, puisqu’il est fait état d’une très faible présence de mineurs.

De même, il conviendrait de distinguer les courses de taureaux avec ou sans mise à mort, là où le texte, de manière peu subtile, prévoit une interdiction globale.

Sur le plan pénal, plusieurs difficultés se posent, à commencer par la question de la responsabilité, qui incomberait de manière disproportionnée à l’organisateur de l’événement en cas de présence d’un mineur. Qu’en est il du jeune qui aurait enfreint la loi et de ses parents ? outre, la présence d’un mineur aurait pour conséquence de requalifier les corridas et les combats de coqs en sévices graves envers les animaux, entraînant de fait de lourdes peines et ouvrant la voie à une interdiction de principe. Cela n’est tout simplement pas

Par ailleurs, au delà de la problématique de la responsabilité des parents, se pose la question de leur appréciation, puisqu’une telle interdiction limiterait l’exercice de l’autorité parentale.

territoires ultramarins où la tradition des combats de coqs est encore très implantée. Le Sénat, chambre des territoires, enverrait alors un message totalement en décalage par rapport à ce qu’il tente toujours de faire : privilégier le dialogue et la concertation locale.

pas de modification du code pénal. Je terminerai en saluant le travail précis et éclairant de notre collègue Louis Vogel. Sa mission n’était pas aisée, mais il a su trouver les arguments aussi bien juridiques que politiques pour nous démontrer le caractère inopportun de la proposition de loi. Pour l’ensemble de ces raisons, les

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, spectacle culturel pour certains, infâme torture pour d’autres, la corrida et les combats de coqs sont de ces sujets qui font débat, parfois jusque tard dans la nuit,

peuvent assister à une corrida, dont le droit ne nie pas qu’elle constitue un acte de maltraitance et de cruauté, mais le tolère au nom de la tradition. insiste, alors qu’une disposition protège les enfants de l’exposition à la violence, une autre, qui ne réfute pas la violence de la corrida, la permet. Comment accepter cette contradiction ? D’autres pays, comme l’Équateur, ont fait un choix clair en interdisant les corridas aux mineurs, se conformant ainsi aux recommandations du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, qui s’est dit « préoccupé par l’état de santé mentale des enfants exposés à la violence de la tauromachie ». En 2016, le même comité demandait à la France de « redoubler d’efforts pour faire évoluer les traditions et les pratiques violentes qui ont un effet préjudiciable sur le bien être des enfants, et notamment d’interdire l’accès des enfants aux spectacles de tauromachie

par leurs proches. Des études, comme celle de l’université de Madrid en 2009, montrent clairement que la majorité des enfants réprouvent spontanément la corrida.

entraîne, selon les études, une perturbation des valeurs, une diminution de l’empathie et une fragilisation du sens moral, qui peuvent les pousser à réaliser eux mêmes des actes répréhensibles envers les animaux ou même les humains. Des études ont ainsi démontré que « le fait d’être témoin de maltraitance animale est un facteur prédictif […] pour […] le harcèlement scolaire chez les enfants Allons nous continuer d’ignorer ces éléments, bien documentés, et le droit pénal sous le seul prétexte de l’existence de traditions ? La protection de l’enfance repose sur le fait, avéré, que l’exposition à des actes de violence contrevient au bon développement de l’enfant. Il n’est plus acceptable que la corrida, dont la seule justification légale est d’être une tradition ininterrompue, échappe à l’ensemble des prescriptions morales et juridiques de la protection de l’enfance : celle ci doit pouvoir s’appliquer

J’ai salué, en commission, le grand talent d’équilibriste de notre collègue Louis Vogel, qui a trouvé des arguments juridiques

Je me permettrai de parler également des combats de coq, mais de manière moins enflammée, même si, au fond, le raisonnement est le même. Vous n’en avez jamais vu ! Pour ma part, je voterai ce texte, mais je souhaite présenter les arguments de mes collègues, dont certains sont présents et s’exprimeront sans doute tout à l’heure, qui s’opposent à cette proposition de loi.

Après tout, les ordalies et l’écartèlement ont été des traditions judiciaires : on peut se féliciter qu’elles n’aient pas été préservées. Même la pensée conservatrice, dont je ne me réclame pas à titre personnel, sépare le bon grain de l’ivraie et ne voit pas dans toute tradition une sainte chose incontestable.

juridiquement contestable, comme l’a brillamment démontré notre rapporteur, est perçue comme un texte d’abolition de la corrida et des combats de coqs. Même si je respecte la liberté des groupes et si j’ai de la considération pour l’auteure de la proposition de loi,

dans un contexte politique, économique et social où le bloc parlementaire central doit faire face à l’activisme des extrêmes, lesquels n’ont qu’un seul but : celui de paralyser le fonctionnement normal de la Nation et de ses institutions.

Laissons donc aux parents le droit sacré d’exercer leur autorité parentale et de juger si leurs enfants peuvent les accompagner aux arènes pour assister à une corrida, organisée dans le cadre juridique dérogatoire qui reconnaît cette tradition comme un patrimoine culturel immatériel. Ne détruisons pas, par l’adoption de cette proposition de loi, la pratique de la tauromachie, qui irrigue toute une culture populaire dans nos territoires, entre la région des Garrigues et la Méditerranée, entre les Pyrénées et la Gascogne.

de plateformes pornographiques dans la manière dont ils empêchaient, ou pas, les mineurs d’accéder à leurs sites. C’est bien la société qui doit fixer les limites : on ne se réfugie pas derrière l’autorité parentale

Au fond, la question qui nous est posée est simple : peut on, sans risque pour la sécurité psychique de l’enfant, l’exposer à un spectacle répété d’actes de cruauté et de sévices graves conduisant à la mort d’un animal ? Je ne reviens pas sur tous les éléments qui ont été évoqués, la réponse est clairement non. On ne peut pas accepter de

Le scrutin est clos.

loi. Rien ne justifie que l’on autorise, voire que l’on incite, un enfant à tuer un animal de façon gratuite, à enfoncer plusieurs fois dans l’échine d’un veau son épée ou ses banderilles, jusqu’à le poignarder dans la nuque pour l’achever. Cela mérite t

Quel est l’avis de la commission ?

L’amendement de Mme Poncet Monge ne nous avait pas paru nécessaire. En effet, dans le texte que nous défendions, les écoles taurines sont bien évidemment visées. Pourquoi ?

Sur ce point, je suis d’accord avec mon collègue et ami Arnaud Bazin. Je pense en effet que le texte que nous examinons mettait en péril, même sans l’amendement de Mme Poncet Monge, les écoles taurines. Je ne doute pas des

Assemblée. Mes chers collègues, je vous rappelle que, si ces amendements de suppression étaient adoptés, il n’y aurait plus lieu de voter sur l’ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les deux articles qui la composent auraient été supprimés. Aucune explication de vote sur l’ensemble

La remarque de Laurent Burgoa vis à vis du président Patriat était tout à fait cordiale, amicale et sympathique. Un peu d’humour n’empêche pas des débats sérieux

vote. Je respecte toutes les positions et comprends très bien que tout le monde n’apprécie pas

Le scrutin est clos.